dans notre texte doivent contribuer au développement d'une stratégie qui assure la résilience alimentaire de nos territoires tout en l'articulant avec la sécurité nationale.

champ de la responsabilité des élus, s'agissant de pourvoir à l'alimentation de nos concitoyens, compétence trop longtemps oubliée en raison de la prospérité de nos sociétés dépendantes du pétrole. Je tiens à souligner que le texte soumis aujourd'hui à notre assemblée fait écho au travail mené par Stéphane Linou, pionnier du mouvement locavore en France et ancien conseiller général de l'Aude.

Il a récemment mené une enquête auprès de différentes personnalités et institutions sur les rapports entre ordre public et non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaires, dont il a récemment publié les conclusions sous le titre : « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». Le résultat de cette étude est édifiant : nous sommes confrontés à un risque réel, mais celui-ci n'a jamais été envisagé en tant que tel, et encore moins évalué. En effet, alors que, au fil des scandales sanitaires survenus ces dernières années, le « bien manger » s'est imposé comme enjeu de santé publique, un pan entier du sujet n'est jamais évoqué : celui de l'articulation entre l'ordre public et la continuité alimentaire. Par le passé, garantir les conditions d'une sécurité alimentaire minimale était un pilier de la légitimité politique des élus. Il est vrai que notre modèle agricole a longtemps reposé sur une conception du foncier nourricier, s'appuyant sur un aménagement multifonctionnel qui occupait une place stratégique. Aujourd'hui, production et consommation ne sont plus territorialisées ; même les zones rurales sont dépendantes et vulnérables, « alimentairement malades », car elles aussi sont perfusées par le ballet des camions de la grande distribution. À l'heure des cyberattaques, du dérèglement climatique, du délitement du lien social et du terrorisme, la production, la distribution et l'approvisionnement alimentaires ne semblent pas suffisamment analysés en termes de risque stratégique. Il suffit d'une annonce de blocage routier pour que les magasins ou les stations-services soient vidés et deviennent le théâtre d'émeutes, avant même toute pénurie. Force est de constater un déficit avéré s'agissant de notre capacité à subvenir localement à l'un de nos besoins élémentaires, celui de se nourrir à un niveau suffisant en cas d'événement majeur. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'il n'existe pas, à ce sujet, de véritable plan de préparation des populations. Pour l'heure, l'exécutif ne dispose que de réponses ponctuelles d'urgence telles que les plans Orsec, qui ont démontré leur efficacité en cas d'événements exceptionnels, qu'il s'agisse de phénomènes climatiques ou de conflits sociaux.

C'est pourquoi nous formulons six propositions, assez simples à mettre en place, pour commencer à réorganiser plusieurs secteurs de la production, de l'alimentation et de la préparation des populations. Il nous faut d'abord définir une réelle stratégie de territorialisation des productions alimentaires. Pour cela, une révision de certains textes de loi serait urgente- je pense notamment à la loi de modernisation de la sécurité civile et à la loi de programmation militaire.

Autre piste de travail : se doter d'un texte pour protéger, sauver dirais-je même, le foncier agricole, en partenariat avec tous les acteurs de la filière. Un tel texte est attendu avec impatience, tant par les élus que par les agriculteurs eux-mêmes.

la Confédération paysanne, Jeunes agriculteurs, la Coordination rurale et même l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Il s'agit d'inscrire l'environnement, les ressources naturelles et le foncier dans une véritable stratégie de solidarité territoriale. Garantir les conditions d'un niveau minimal de sécurité et d'approvisionnement alimentaires est un devoir pour les autorités. Il y va de leur responsabilité et du lien de confiance qu'elles entretiennent Qu'il s'agisse des élus ou des autorités institutionnelles, les instances décisionnelles devraient s'assurer d'être en mesure de garantir l'existence d'une chaîne résiliente allant du foncier agricole jusqu'au consommateur.

cosignée par l'ensemble des membres du groupe RDSE vise à nous conduire à nous interroger collectivement sur la souveraineté et la sécurité nationales.

Alors que les pouvoirs publics perdent peu à peu la main sur des infrastructures d'intérêt vital, telles que les plateformes aéroportuaires, ou sur la gestion de l'eau, il est essentiel et urgent de se préoccuper de la résilience alimentaire des territoires, pour des raisons évidentes de sécurité nationale. C'est pourquoi, au nom des membres du groupe RDSE, je vous invite à adopter cette proposition de résolution et vous remercie par avance, mes chers collègues, pour votre soutien. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution sur la résilience alimentaire traite d'une question essentielle pour nos territoires, celle de leur autonomie alimentaire, à travers le prisme inédit de la sécurité en cas de situations extrêmes. Nous partageons pleinement le constat dont partent les auteurs de ce texte. En effet, les grands bouleversements climatiques et économiques que nous connaissons imposent de repenser notre modèle de production et de consommation alimentaires.

Il est évident que, face à la récurrence des aléas, climatiques comme économiques, notre agriculture devra être plus résiliente, plus diversifiée. Nous avons plus que jamais le devoir de protéger nos terres agricoles de l'artificialisation.

Il se trouve que les sénateurs du groupe socialiste ont fait de nombreuses propositions, ces dernières années, pour améliorer la résilience de notre agriculture. Outre nos interventions sur les différents textes agricoles ou au moment de la discussion du budget, nous avons déposé plusieurs textes qui ont été examinés en séance publique. premièrement, une proposition de résolution visant à encourager le développement d'outils de gestion de l'aléa économique en agriculture, adoptée le 6 avril 2016. Nous préconisions notamment d'activer le mécanisme de stabilisation des revenus au sein du deuxième pilier de la

une proposition de loi visant à mettre en place des outils de gestion des risques en agriculture, qui a été adoptée le 30 juin 2016. Elle s'inscrivait dans la continuité de la proposition de résolution que je viens de mentionner. Nous proposions de mettre en place des fonds de stabilisation des revenus agricoles dans chaque région, d'expérimenter la mise en oeuvre dans les territoires de mécanismes de gestion mutualisée des risques économiques agricoles,

L'objectif était d'encourager le développement des PSE, entendus comme les externalités positives de l'agriculture, c'est-à-dire l'ensemble des effets positifs susceptibles d'être engendrés par des modes de production ou des pratiques agricoles adaptés. Nous proposions ainsi de rémunérer de façon permanente les pratiques agricoles ayant une plus-value environnementale et La problématique spécifique de la résilience alimentaire, objet de la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui, est une question centrale. Elle est en effet au coeur de nombreux enjeux de résilience de nos territoires, tant environnementaux qu'économiques, sociaux ou sociétaux la réduction des émissions de carbone liées aux transports ; la diminution de la vulnérabilité et de la dépendance aux matières premières importées ; la sécurisation des approvisionnements ; l'amélioration de la qualité et de la traçabilité des produits consommés ; la maîtrise de la consommation individuelle et de la pollution associée ; la relocalisation des emplois sur les territoires ; le développement d'une économie locale plus inclusive qui fasse une place à tous et redonne du sens aux missions fondamentales des agriculteurs locaux, à savoir nourrir le territoire et entretenir ses paysages. Or, en matière d'alimentation, nos territoires ne maîtrisent qu'une part infime des ressources agricoles qui serviront à la consommation de leurs populations. Une étude du cabinet Utopies a ainsi évalué le taux d'autonomie alimentaire des cent premières aires urbaines françaises à seulement

Sur une vaste partie de notre territoire national, il ne manque donc plus que la volonté politique pour organiser la reconnexion entre production et consommation de produits agricoles destinés à l'alimentation. Les territoires à forte densité urbaine ou dont les caractéristiques géographiques limitent le potentiel agricole- Paris, Marseille, Bordeaux, Nice, Montpellier, Creil, Forbach -devront, plus encore que les autres, être accompagnés dans le développement de nouvelles formes d'agriculture urbaine ou semi-urbaine. Nous partons de loin et, pour accroître significativement l'autonomie alimentaire de nos territoires, il faudra la mobilisation de tous- pouvoirs publics nationaux, élus locaux, citoyens -autour d'une prise de conscience partagée des enjeux. À ce titre, je souhaite remercier Françoise Laborde et son groupe : la discussion de la présente proposition de résolution contribue à cette nécessaire prise de conscience. Je voudrais maintenant revenir sur l'angle choisi

Ils proposent d'anticiper une conséquence de la multiplication des aléas climatiques et des crises économiques, qui serait un « angle mort » de nos politiques publiques : le déclenchement de troubles importants de l'ordre public sous forme d'émeutes, de blocages, etc. Cette approche, qui aurait pu être qualifiée de catastrophiste, voire prêter à sourire, il y a quelques années, ne peut

Cela conduit l'auteure principale de cette étude à nous alerter sur le fait que « les chocs climatiques subis par la production agricole contribuent aux pics de prix et à la famine et pourraient déclencher d'autres risques systémiques, comme des troubles politiques ou des migrations Deuxièmement, des chercheurs de l'Institut sur le changement climatique de Potsdam, en Allemagne, mettent en garde contre le risque « multiplié par vingt » de canicules simultanées affectant des zones de l'hémisphère Nord représentant jusqu'à un quart de la production mondiale. Ces canicules plus nombreuses et de plus en plus sévères menacent « la disponibilité en nourriture non seulement dans les régions affectées mais dans des régions plus lointaines qui peuvent enregistrer pénuries et augmentations des prix Les effets critiques des bouleversements climatiques anticipés ne peuvent donc plus être assimilés à des scénarios de science-fiction.

à savoir la reconnaissance de notre agriculture comme secteur d'activité d'importance vitale (SAIV). Cette interrogation ne porte pas sur le bien-fondé de l'intention. Il est évident que la préservation de nos terres et la protection de nos agriculteurs doivent être des priorités nationales. La reconnaissance de la production alimentaire et du foncier agricole nourricier en tant que SAIV ne pose donc pas un problème de fond. Toutefois, en vue de sa mise en oeuvre, cette préconisation nécessiterait une analyse plus fine que celle figurant dans le très court exposé des motifs de la proposition de résolution. Celui-ci laisse en effet un certain nombre de questions en suspens. Concrètement, comment la reconnaissance du foncier agricole en tant que SAIV permettrait-elle de lutter contre l'artificialisation des sols ou l'achat de nos terres par des investisseurs étrangers ? Comment pourrait-elle encourager la relocalisation de nos productions dans les territoires ? Comment seront désignés les opérateurs d'importance vitale parmi la multitude de structures ou d'organisations agricoles ? Quels seront les sites plus particulièrement sensibles désignés points d'importance vitale : les terres d'élevage extensif seront-elles traitées sur le même pied que les grands vignobles, par exemple ? Par ailleurs, il faut rappeler que l'alimentation est déjà reconnue comme un SAIV. Le ministère de l'agriculture a d'ailleurs publié un guide des recommandations pour la protection de la chaîne alimentaire contre les risques d'actions malveillantes, criminelles ou terroristes en 2014. Dans ce cadre, faut-il vraiment envisager la création d'un nouveau SAIV ? Un simple « élargissement » de l'existant ne pourrait-il suffire ? Même si ces interrogations, essentiellement d'ordre technique, restent entières en l'état du texte de la proposition de résolution, nous considérons, avec mes collègues du groupe socialiste et républicain, que les questions fondamentales soulevées méritent d'être très sérieusement prises en compte, non seulement par notre assemblée, mais aussi et surtout par les ministères concernés. C'est pourquoi nous voterons en faveur de l'adoption de cette proposition de résolution. La parole est à M. François Bonhomme. Monsieur le président, monsieur

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution qui nous est soumise cet après-midi met en exergue une réalité qu'aucun d'entre nous ne saurait contester.

Il est évidemment de la responsabilité de l'État de prendre en compte cette situation afin d'assurer une meilleure protection de nos agriculteurs, mais aussi de la population. De ce point de vue, l'État a très largement échoué à assumer pleinement ce rôle de prévention qui lui revient. Dans cette optique, le récent rapport d'information de nos collègues Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart rappelait que l'État a ponctionné le fonds de prévention des risques naturels et majeurs. Les communes constituent le premier échelon de prévention des catastrophes naturelles. Pourtant, dans leur rapport relatif à la gestion des catastrophes naturelles dans les outre-mer, nos collègues Mathieu Darnaud, Victoire Jasmin et Guillaume Arnell soulignaient que, à ce jour, seules trois

afin d'apporter des réponses concrètes à la menace de la survenance de catastrophes climatiques majeures. Certes, les plans Orsec permettent à l'État de répondre à ces situations d'urgence et leur efficacité a été prouvée. Mais celle-ci dépend aussi de la capacité des communes à anticiper la survenance de pareils événements. Dès lors, je ne peux qu'être sceptique à l'égard de cette proposition de résolution qui, à mon sens, fait l'impasse sur les plans de prévention déjà en place et repose sur l'hypothèse que l'État ne serait pas capable de gérer des situations de crise. Par ailleurs, cette proposition de résolution relève d'une vision ultra-collectiviste de l'agriculture française, en prévoyant une forme de collectivisation au bénéfice de l'État de terres agricoles et des ressources qui leur sont

Permettez-moi enfin de rappeler le mouvement de démocratisation de la consommation d'aliments issus de l'agriculture biologique. À ce titre, le cap des 2 millions d'hectares cultivés en agriculture biologique a été franchi.

C'est la première fois, en effet, que le Sénat se saisit de la question de la résilience alimentaire. Le sujet n'est pourtant pas nouveau. Depuis plusieurs décennies, la communauté scientifique nous alerte sur les risques que le réchauffement climatique fait peser sur nos systèmes de production et de consommation ; nous y reviendrons. La question occupe par ailleurs une place de plus en plus importante dans le débat public. Au-delà de l'enjeu purement alimentaire, c'est la résilience même de nos sociétés face aux crises environnementales, économiques ou politiques qui est en cause. La littérature sur ce sujet est foisonnante ; je ne m'y attarderai pas.

parlementaires. Ses auteurs entendent alerter le Gouvernement sur notre vulnérabilité alimentaire et sécuritaire en cas d'événements de force majeure. Ils proposent de mettre en place une stratégie de « territorialisation » des productions alimentaires, d'établir une cartographie des flux de production et de développer une culture du risque. Ils entendent, par ailleurs, inciter le Gouvernement à présenter un projet de loi de sauvegarde du foncier agricole, à engager une révision de la loi de programmation militaire et à intégrer la notion de résilience alimentaire des territoires dans la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Force est de constater, mes chers collègues, que l'actualité de ces dernières années leur donne en grande partie raison. En août 2019, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat s'est ainsi penché sur la question de la sécurité alimentaire dans son rapport spécial consacré aux terres émergées. Ce rapport souligne notamment que le changement climatique a une incidence sur les quatre piliers de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité des produits agricoles, l'accès à la nourriture, l'utilisation qui en est faite et la stabilité de l'approvisionnement. Ces dernières années, la résilience des systèmes alimentaires a par ailleurs occupé une place centrale dans la stratégie des institutions et des ONG d'aide aux aux populations les plus démunies. La répartition géographique de celles-ci coïncide, en effet, avec la carte des régions du monde le plus durement affectées par le changement climatique. Les périodes de sécheresse, combinées à un fort accroissement du nombre et de la gravité des catastrophes naturelles, augmentent leur vulnérabilité face aux pénuries alimentaires. La récurrence des crises dans le monde a ainsi mis en lumière la nécessité de faire porter la réflexion sur l'urgence et le développement. et le développement. L'aide humanitaire ne préparant que rarement les populations aux crises futures, il est nécessaire de traiter la question de la sécurité alimentaire de manière plus intégrée et durable. Les risques pesant sur la sécurité alimentaire ne s'arrêtent toutefois pas aux frontières des pays défavorisés. La France, comme l'ensemble des pays industrialisés, est elle aussi directement concernée, malgré une production de denrées agricoles importante et supérieure à ses besoins. La réduction des surfaces agricoles, l'artificialisation des terres, la raréfaction des ressources hydriques, l'hyper-sophistication des chaînes d'approvisionnement et la dépendance extrême aux énergies fossiles sont autant de facteurs de facteurs qui rendent notre système alimentaire particulièrement vulnérable face aux menaces systémiques. Cette vulnérabilité est exacerbée dans les territoires d'outre-mer, en raison de leur isolement et de leur insularité. Ces dernières années, ces territoires ont été confrontés à des crises naturelles et politiques qui ont affecté parfois durablement leur approvisionnement. Permettez-moi de m'y attarder un instant. En septembre 2017, l'ouragan Irma a frappé de plein fouet les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, provoquant des difficultés d'accès aux produits de première nécessité dans les heures et les jours qui ont suivi la catastrophe. Le manque d'organisation et de réserves de nourriture a été à l'origine de scènes de violences et de pillages. En mai 2018, la Désirade et de Terre-de-Bas, en Guadeloupe, ont vu leurs ports bloqués par l'arrivée d'immenses radeaux d'algues sargasses, les coupant presque entièrement du monde. Si le phénomène n'est pas ancien, il devrait s'accentuer dans les années à venir. En décembre 2018, l'île de la Réunion a connu elle aussi une rupture d'approvisionnement en biens de première nécessité en raison du mouvement des « gilets jaunes ». Près d'un millier de conteneurs renfermant des produits frais, des matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux ou des médicaments et du matériel médical sont ainsi restés en attente de livraison. Ces situations sont d'autant plus problématiques que les territoires d'outre-mer connaissent une dépendance croissante aux importations. Tous territoires confondus, les marchandises produites localement ne représentent que le quart des marchandises vendues par les distributeurs. Près de 95 % de ces marchandises sont d'ailleurs acheminées par voie maritime. Ces importations agroalimentaires sont rendues nécessaires par l'insuffisance de la production locale, malgré la mise en place de régimes d'aide. Il est donc, là aussi, nécessaire d'encourager davantage le développement des filières de diversification. Compte tenu de ces éléments, notre groupe votera en faveur de l'adoption de cette

La succession d'événements climatiques extrêmes, les rapports successifs du GIEC, tout comme ceux du Haut Conseil pour le climat et de toutes les instances chargées de mesurer les effets de l'action humaine sur le climat, ainsi que l'impératif de réduire nos émissions de gaz à effet serre, l'exploitation irrationnelle de ressources naturelles finies : tout cela peut susciter un sentiment de désespoir, de colère, de sidération, voire de dépression, mais aussi, chez certains, un déni de la réalité du changement climatique, tant les défis environnementaux et économiques auxquels nous sommes confrontés sont redoutables. L'urgence n'a sans doute jamais aussi prégnante

Or nous pouvons encore agir ! Des centaines de milliers de personnes marchent pour le climat ; des milliers de jeunes se mobilisent ; on voit partout émerger d'autres manières de vivre, des propositions pour promouvoir un mode de vie respectueux de la planète. C'est pourquoi, si nous partageons le point d'arrivée de la proposition de résolution du groupe RDSE, nous n'en approuvons pas les préconisations. En matière agricole, cela fait des années que l'obsession de l'accroissement de la productivité a pris le pas sur toute autre considération et a provoqué la disparition massive des petites exploitations, jugées moins rentables et moins capables de faire face au défi de la concurrence, notamment dans le cadre d'une libéralisation des marchés agricoles. Pour notre part, nous avons toujours défendu l'idée que seule une agriculture à visage humain, une agriculture locale et paysanne permettra de relever les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Cela fait des années que nous défendons une agriculture familiale, locale, permettant une production de qualité, un « réinvestissement » des campagnes et une transition écologique, ayant pour objectifs la souveraineté alimentaire et une rémunération juste pour celles et ceux qui travaillent la terre. Pour cela, il faut une relocalisation de la production afin de privilégier les circuits courts, qui permettent une meilleure traçabilité des produits et favorisent de nouvelles formes de distribution. Il faut un assouplissement du code des marchés publics, par exemple

mise en oeuvre permettrait d'éviter une fracture territoriale et sociale en matière d'accès à une alimentation de qualité. Dans le même ordre d'idées, il est impératif de s'opposer aux traités de libre-échange,

ce même libéralisme qui fait le départ entre, d'un côté, ceux qui pourront monter en gamme, et, de l'autre, la majeure partie des gens, ceux qui devront acheter à manger au prix le plus bas, dans les conditions environnementales les plus sévères. Malgré ces réserves, nous soutenons l'initiative des auteurs de la proposition de résolution. Si la peur ne peut être un moteur, il n'en demeure pas moins que les questions soulevées et l'invitation faite au Gouvernement d'amorcer un changement radical en matière agricole sont pertinentes. la résilience alimentaire doit devenir un sujet prioritaire dans l'agenda politique, pour que les élus, les experts en sécurité et en gestion de risques, les représentants de la production et de la distribution alimentaires s'en emparent et pour qu'une stratégie de prévention et un plan de résilience soient élaborés afin de prévenir le risque de pénurie. Oui, la dissociation entre les territoires où sont produits les aliments et ceux où ils sont consommés constitue un risque réel. Il est indispensable de le prendre en compte dans la et dans les plans de gestion des risques. Non, le foncier agricole n'est pas sécurisé par un corpus législatif le protégeant de l'accaparement par des puissances étrangères. En outre, l'artificialisation des terres réduit les surfaces agricoles. Dès lors, relocaliser la production, accélérer le passage à l'agriculture biologique, privilégier les circuits courts, cartographier tous les producteurs, évaluer différentes possibilités en matière de transport et de distribution

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pas une année ne passe sans que nous ne recevions des images venues d'ailleurs montrant les désastres de la faim. La faim frappe presque toujours les pays meurtris par les conflits et les guerres. Elle en constitue bien souvent l'une des conséquences malheureuses. La faim se trouve aussi à la source de nombreuses tensions qui déchirent les sociétés et ébranlent les régimes politiques.

qui nourrit les Français et exporte ses denrées en Europe et dans le monde. Tel est aujourd'hui le véritable fondement de notre résilience alimentaire. Il ne faut donc pas se tromper de combat. L'agriculture française, la première d'Europe, est aussi l'une des plus diversifiées au monde.

Cette proposition de résolution, même si elle nourrit un discours trop alarmiste fondé sur un constat quasiment apocalyptique, a le mérite d'attirer notre attention sur cette problématique. C'est l'occasion de mettre en relief ce qui nous semble essentiel pour véritablement garantir notre autonomie et notre souveraineté alimentaires. Cette problématique n'est pas nouvelle, mais elle se présente aujourd'hui sous un jour inédit, notamment en raison de l'effet combiné de la mondialisation des échanges et du dérèglement climatique. Ces deux tendances transformeront encore à l'avenir nos modes de production agricole, ainsi que nos habitudes de consommation. C'est dans ce cadre que nous devons proposer une vision ambitieuse et pragmatique de la résilience alimentaire. Cependant, cette vision ne doit pas se développer au gré des tendances consuméristes et au mépris de notre passé, notamment de notre passé récent. Il n'y a pas si longtemps encore, tout particulièrement au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France souffrait massivement de la faim. Notre pays est parvenu à l'éradiquer ; c'était d'ailleurs un objectif fondateur de l'Union européenne, qui

pas, l'agriculture a très rapidement constitué un pilier essentiel de la construction européenne ! Il ne s'agit pas de nier les défis auxquels notre modèle agricole devra faire face dans le futur. Il s'agit seulement de se souvenir d'où l'on vient pour bien comprendre où l'on veut aller. Aujourd'hui, notre pays a toutes les raisons d'être fier de son agriculture. La France est le premier producteur agricole européen, devant l'Allemagne et l'Italie. Alors que notre pays affiche malheureusement, depuis plusieurs années, un déficit commercial structurel, notre industrie agroalimentaire présente, elle, un excédent structurel. France se trouve d'ores et déjà en situation d'autosuffisance alimentaire. Elle concourt également à l'autosuffisance de l'Europe et contribue à alimenter le marché mondial, ce qu'elle doit continuer à faire. Certes, l'autosuffisance n'implique pas nécessairement la résilience,

Si nous avons conquis notre indépendance alimentaire, c'est d'abord par le développement de nos capacités de production et des échanges commerciaux avec nos partenaires européens.

Notre production nationale tend à stagner, notre rang dans les échanges internationaux se détériore et la place qu'occupent les importations dans notre alimentation augmente, comme l'a mis en exergue un récent débat au Sénat.

Alors que notre planète devrait compter 10 milliards d'êtres humains en 2050, notre capacité collective à nourrir tout ce monde est incertaine. Si notre agriculture est à à la pointe en matière environnementale et figure parmi les plus durables au monde, elle peut encore réaliser d'importants progrès en termes de productivité, en misant sur l'innovation. Dans cette optique, toutes les évolutions sociétales qui concourent à soutenir une agriculture nationale, et donc locale, vont dans le bon sens. Le développement des circuits courts ou la transition de notre agriculture participent d'une politique agricole ambitieuse. Nous ne souhaitons aucunement opposer les modèles ; au contraire, il faut les rendre complémentaires et les combiner. La résilience alimentaire

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à remercier Françoise Laborde, dont l'initiative nous permet d'échanger sur ce sujet fondamental de notre quotidien : notre alimentation. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui a pour objet de remettre au centre du débat la question de la résilience alimentaire et de la capacité de nos territoires à faire face à des crises profondes et durables.

La raréfaction des terrains, notamment aux abords des villes, en fait une ressource convoitée qu'il faut préserver, par exemple contre les appétits de puissances étrangères. Par ailleurs, l'agriculture de proximité et le développement des circuits courts sont une source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs.

Certaines préconisations de cette proposition de résolution semblent de nature à imposer de nouvelles contraintes à des agriculteurs déjà assujettis à de nombreux impératifs. Appuyons-nous plutôt sur les dizaines de solutions agroécologiques qu'ils nous proposent

Enfin, j'observe une certaine contradiction entre une localisation stricte des productions et le défi de nourrir 10 milliards d'habitants ! En tant qu'élus des territoires, nous devons veiller à ce que les textes que nous votons prennent la mesure des difficultés actuelles des agriculteurs,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de résolution de notre collègue Françoise Laborde sur la résilience alimentaire des territoires et la sécurité nationale. la sécurité nationale. Ce texte trouve son origine dans un mémoire de recherche intitulé « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». Il s'agit d'une enquête menée au sein des milieux de la défense, de l'agriculture, de la sécurité et de l'alimentation, dont l'auteur analyse un impensé : la France est-elle préparée à une pénurie alimentaire ?

J'estime qu'elle décrit un risque dont la probabilité n'est pas démontrée. En cas de catastrophes naturelles, la chaîne d'approvisionnement est déjà prise en compte dans le cadre des plans Orsec, qui s'appuient sur la préparation commune de tous les acteurs publics et privés. L'ensemble est coordonné par le préfet. Le plan Orsec permet de faire face à tous types de situations d'urgence, de protéger les populations, l'environnement et les biens. Il est mis à jour par par l'actualisation des bases de données réalisée par chacune des personnes publiques et privées, conformément à l'article R. 741-6 du code de la sécurité intérieure. En outre, cette proposition de résolution dénonce « la logique de marché qui ignore la sécurisation du foncier agricole nourricier ». Est-ce à dire qu'il faudrait envisager la collectivisation des terres agricoles afin de protéger les populations ? Cela a déjà existé à l'époque de Staline, sans empêcher d'ailleurs des famines ... La question du foncier agricole est complexe et mérite mieux que des postures idéologiques éloignées du quotidien des agriculteurs. Les outils de protection et de régulation du foncier agricole sont élaborés aux fins de préserver les exploitations agricoles dans le respect du droit de propriété. la proposition de résolution affirment ensuite que « le foncier agricole n'est pas sécurisé par un corpus législatif qui protège nos terres nourricières de l'accaparement par des puissances étrangères Je rappelle que la loi du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres et au développement du biocontrôle a instauré un dispositif législatif tendant à renforcer la transparence des acquisitions du foncier agricole par les sociétés, en les obligeant à s'appuyer sur une société dédiée au portage du foncier pour toute nouvelle acquisition ou tout apport de foncier. La transparence de ces opérations est ainsi assurée. Pour construire des solutions qui répondent aux besoins des agriculteurs en matière de foncier agricole, il est préférable d'être à l'écoute des agriculteurs sans les stigmatiser. L'évolution du foncier agricole doit se construire avec les agriculteurs, et non contre eux. de la proposition de résolution observent avec raison que les agriculteurs exploitent ou utilisent des installations indispensables à la vie de la Nation, mais soulignent qu'ils ne sont pas considérés comme des opérateurs d'importance vitale. des opérateurs d'importance vitale. Ceux-ci sont désignés, pour chaque secteur d'activité d'importance vitale, par arrêté. Ils ont pour obligation d'analyser les risques, d'établir un plan de sécurité prenant en compte les attendus de la directive nationale de sécurité au titre de laquelle ils ont été désignés désignés et d'identifier leurs points d'importance vitale, qui feront l'objet d'un plan particulier de protection à leur charge et d'un plan de protection externe à la charge du préfet de département. Rappelons que les agriculteurs ont toujours joué un rôle vital pour les populations et l'économie de notre pays sans qu'il soit nécessaire de les considérer comme des opérateurs d'importance vitale.

qu'il faille changer de système et mettre les agriculteurs sous la tutelle de l'État. Je ne voterai pas cette proposition de résolution qui instrumentalise les peurs et ne se fonde sur aucune démonstration probante. La parole

La production locale agricole demeure essentielle à la vie et appartient au patrimoine français » : nous sommes d'accord. « La planète comptera 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050, il est donc primordial de préserver les terres arables » : nous La logique de marché menace la sécurisation du foncier agricole nourricier » : nous sommes d'accord. « L'environnement et les ressources sont des biens qui doivent être gérés dans une véritable stratégie de solidarité territoriale L'excellent rapport de nos collègues Ronan Dantec et Jean Yves Roux fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective nous a tous ébranlés : oui, le changement climatique est là, il n'est pas pour demain. L'agriculture doit évoluer. Les ressources hydriques doivent être gérées autrement, il faut désormais s'organiser collectivement pour parer aux pénuries d'eau. L'ensemble de nos pratiques doivent être adaptées. Nous devons collectivement nous préparer à des situations extrêmes et à des événements climatiques exceptionnels.

De même, la perspective d'une révision de la loi de programmation militaire pour intégrer la production et le foncier agricoles comme secteurs d'activité d'importance vitale suscite les plus vives inquiétudes dans le monde rural, qui anticipe toutes les lourdeurs et complications supplémentaires qui pourraient en découler.

Les ministères de l'intérieur et de la défense ont-ils été consultés sur ce point, car ils seraient en première ligne de ces éventuelles réorganisations ? L'instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d'importance vitale prévoit bien le point clé suivant La constitution d'une zone d'importance vitale doit apporter une plus-value opérationnelle. » Est-ce le bon outil pour éviter « le risque d'accaparement par des puissances étrangères »

Tout le monde nous vante les vertus des circuits courts, mais moi, je produis de quoi nourrir 1 000 personnes, et j'habite un village de 200 habitants. » Les choses ne sont donc pas si simples. Même si le ballet des camions de la grande distribution apparaît comme une aberration environnementale, les comportements du consommateur ont changé. Les circuits courts ont leurs limites et ne peuvent être la solution universelle. Les marchés agricoles sont mondiaux, et si la « territorialisation des productions alimentaires » est un concept rassurant, elle n'est pas toujours possible. Quelqu'un faisait remarquer ce matin qu'il faudrait alors oublier l'idée de boire du café

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'échéance de 2050, il faudra nourrir 10 milliards de personnes dans un contexte de réchauffement climatique qui va accentuer la pression sur les terres agricoles. Seuls les pays qui auront su préserver leur agriculture de la pression foncière et des aléas climatiques seront en mesure de répondre à la demande mondiale. La France, puissance agricole de premier plan, en est-elle seulement encore capable ? Peut-elle encore aujourd'hui assurer son indépendance alimentaire ? Ce sont les questions que soulève cette proposition de résolution, qui vise à alerter l'exécutif « sur l'importance d'une prise en compte de la territorialisation de la production, de la transformation et de la distribution alimentaires Elle rappelle aussi que les autorités publiques doivent être en mesure de « garantir les conditions d'un niveau minimum de sécurité et d'approvisionnement alimentaire ». Il est en effet de la responsabilité de l'État de garantir notre souveraineté alimentaire, que le général de Gaulle qualifiait d'ailleurs d'« ardente obligation ». Souveraineté alimentaire et autonomie stratégique militaire sont liées. Trouvez-vous d'ailleurs normal, monsieur le ministre, que l'économat des armées françaises ne s'approvisionne pas uniquement avec des produits agricoles français ? Soutien aux armées, soutien aux agriculteurs ! Ces agriculteurs, qui affrontent tellement de difficultés et qui travaillent sans relâche, ne pourront supporter très longtemps l'absence de mesures concrètes pour améliorer leur situation. Le défi qui nous attend consiste à redonner un équilibre à la mondialisation. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas su prendre la mesure de l'évolution de celle-ci. Nous avons appliqué des normes plutôt que de définir une stratégie, et, dans certains secteurs, comme l'agriculture, nous nous sommes retrouvés en compétition avec des concurrents qui ne respectent aucune des règles imposées ; nous avons perdu des batailles.

En plus de mettre en péril la sécurité sanitaire de nos concitoyens, ce phénomène autorise une concurrence déloyale au détriment de nos producteurs. Si rien n'est fait, cette tendance va s'accentuer. Je rappelle que les notions d'autosuffisance et de sécurité alimentaires, qui tiennent aux besoins les plus fondamentaux de la personne, doivent être au coeur de toute vraie politique agricole. Plus que d'une « stratégie de territorialisation des productions alimentaires, d'une cartographie des flux de production alimentaire et d'une préparation des populations » ou « d'une loi de sauvegarde du foncier agricole », comme le prévoit la proposition

Le Gouvernement n'est certes pas responsable de ce dont il a hérité, mais il l'est, en revanche, de ce qu'il a ou non entrepris. Il a fait adopter la loi Égalim, qui a suscité un immense espoir chez les agriculteurs.

Les agriculteurs ont besoin de solutions pérennes, concrètes, immédiates. Il n'y a aucune raison que l'agriculture française ne se redresse pas. Il le faut, c'est un impératif pour notre pays. Je fais partie de ces élus qui pensent que la France a une grande vocation agricole et que notre souveraineté est garantie pour autant que notre autosuffisance alimentaire soit assurée. Notre pays

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte dont nous discutons aujourd'hui aborde une thématique essentielle, puisqu'il traite d'un enjeu de sécurité nationale : la résilience alimentaire.

La sécurité alimentaire est un enjeu de premier plan. Historiquement à la base de l'action publique et de l'ordre public, son importance pour la sécurité civile est aujourd'hui oubliée. Pourtant, dans un contexte marqué par des aléas climatiques de plus en plus nombreux et graves, par des pénuries d'eau inquiétantes, par des prix fluctuants de l'énergie, cette question semble plus que jamais d'actualité. Françoise Laborde a déjà cité, très justement, les nombreux rapports sénatoriaux mettant en avant la nécessité d'anticiper les risques qui pèsent sur notre production alimentaire. Face à ces menaces, nos villes, comme nos campagnes, ne sont pas préparées. En effet, elles sont sous perfusion des grandes surfaces et de leurs systèmes logistiques. Leur taux d'autonomie alimentaire est particulièrement faible : de l'ordre de 2 % pour les aires urbaines, et guère plus pour

la question des outre-mer est ici particulièrement prégnante, puisqu'une part très importante de leur alimentation est importée, depuis des territoires éloignés et des circuits d'approvisionnement vulnérables aux événements climatiques. Face à ces menaces, les pouvoirs publics manquent de réponses : les plans Orsec, prévus pour gérer des crises exceptionnelles et de courte durée, sont insuffisants pour faire face à des aléas climatiques ou à des pénuries de plus long terme.

Des militaires et de nombreuses personnes, au sein des services de l'État et des collectivités locales, se sont montrés très intéressés par son travail. Pour remédier à cette carence, la proposition de résolution comporte des recommandations pertinentes et de bon sens préparation des populations, intégration du lien entre les questions militaires, de sécurité et alimentaires, notamment l'ajout de la production alimentaire et du foncier agricole à la liste des secteurs d'importance vitale pour notre pays.

Pour assurer la résilience des territoires, il faut toutefois aller aujourd'hui plus loin, comme le souligne le texte, qui prévoit d'agir sur le foncier et de favoriser le développement local de systèmes agricole et alimentaire résilients. Les pistes proposées entrent en forte résonance

J'espère que la loi foncière promise par le Gouvernement sera prochainement annoncée. Enfin, l'Association française pour l'étude du sol organisait à Vannes, la semaine dernière, un colloque sur l'érosion des sols, afin de définir des solutions locales et territoriales.

plus, de l'aléa qui fait tout basculer, d'un endettement qui étouffe la vie de l'exploitant et de sa famille, de la peur de recevoir une énième lettre de mise en demeure avant saisie ou de se voir agresser par des associations, mais aussi celui de la perte d'humanité d'une administration devenue frileuse et qui gère des dossiers avant de parler à des femmes et à des hommes. Lentement arrive le burn-out, sujet tabou de notre société. Le suicide en agriculture, c'est tout cela. Alors que faire, tellement la tâche est lourde ? Par quel bout prendre ce fléau ? La loi Égalim avait cerné le coeur du problème : le partage de la valeur, la nécessité d'un juste prix, à la hauteur des heures de travail et des frais de production.

Vous le savez, je ne suis jamais intervenu sur l'agriculture dans cet hémicycle sans aborder ce sujet. Je glisse toujours cette phrase : « et pendant ce temps, un agriculteur se suicide tous les deux jours » ; mais aujourd'hui, c'est un agriculteur tous

Engagés pour défendre les paysans, ils sont venus débattre avec nous, mercredi dernier, comme ils l'avaient fait à l'Assemblée nationale et comme ils le feront au Parlement européen, à Bruxelles. Pour comprendre ce phénomène, j'ai écouté et j'ai lu les messages d'épouses ou de membres de la famille, reçus sur ma boîte aux

Séverine s'inquiète : « En mars 2018, mon frère a tenté de mettre fin à ses jours. Depuis, que de douleurs pour toute la famille : inquiétude, doute et peur ... C'est un homme courageux qui ne peut vivre de son travail. Et je sais ce dont je vous parle, car ma soeur et moi avons repris toute l'administration de son exploitation : trop de papiers à faire ; des délais, des dates et des larmes Sylvie et Pascal m'indiquent : « Le problème du suicide en agriculture est tabou, les témoignages rares. Une libération de la parole réduirait sensiblement le problème. L'administration a un grand rôle à jouer ; qu'elle remette de l'humain dans ses relations avec les paysans. L'agribashing est aussi administratif. » Pascale témoigne : « Femme d'agriculteur depuis plus de vingt ans, j'espère que vous arriverez à faire changer les choses. Mon mari n'a encore jamais sauté le pas, mais j'ai passé des soirées à avoir peur qu'il ne revienne. Je prenais mon téléphone ; s'il ne répondait pas, je recommençais. Je pense qu'il ne s'est jamais douté de mes peurs, mais elles sont bien là et on est impuissant face à ce mal-être. dont l'exploitation est en redressement judiciaire, s'indigne : « Il serait bien que cette loi porte le nom de M. Bergeon, ou de sa femme ou de ses enfants, car ce qu'il faut dire, c'est que la famille est à bout de porter les devoirs, les factures, la comptabilité, les enfants, la maison, son propre travail ... Et tout le monde survit. survit. » Mes chers collègues, je pense que ces quelques témoignages- le ministère en tient des dizaines à votre disposition -posent mieux que de grands discours le problème de fond : la non-rémunération.

j'ai choisi d'inscrire les banques au dispositif de prévention, car je reste persuadé qu'elles ont un rôle majeur à jouer : elles sont au premier plan pour voir les comptes d'exploitation, mais aussi les comptes privés, virer au rouge. Alors, on me rétorque que c'est trop compliqué, qu'on ne peut responsabiliser, par la loi, des personnels déjà soumis à des objectifs et à des procédures de qualité, qu'on ne peut confier cette mission de vigilance à un seul partenaire, que le problème économique n'est pas le seul,

J'ai interpellé des conseillers juridiques, des agriculteurs ; tous relèvent une contradiction : comment peut-on demander à un organisme d'être à la fois celui qui prélève les cotisations sociales, souvent sans ménagements, et celui qui doit vous aider quand ça va mal ? Celui qui montre le bâton et celui qui vous tend la main ?

sur un geste que certains taisent, préférant la version de l'accident du travail, qui ouvre des droits. Il reste désormais à travailler pour trouver des solutions, d'autres solutions. Pourquoi continuer à énumérer les outils, alors que l'on constate leur manque d'efficience ?

avec un objectif essentiel : comment introduire plus d'humanité dans les démarches administratives et les contrôles ? C'est tout un système social qui doit-être réformé. Le combat pour une vie meilleure pour nos agriculteurs doit être mené parallèlement au travers de toutes les actions nationales et européennes. Pour ce faire, nos échanges ne devront pas être clivés par des convictions politiques ; la vie de milliers de paysans en dépend, et on ne peut plus, face à un constat dramatique, en rester à des postures tranchées, qui nient le désarroi des agriculteurs et font offense à la souffrance paysanne. n'avons plus le temps de croiser le fer en opposant les agricultures : conventionnelle, bio, à haute valeur environnementale, raisonnée, à circuit court ... Je vois d'ailleurs avec inquiétude les syndicats s'opposer dans un débat stérile sur l'agri-bashing.

mettre autour d'une même table les banques, la MSA, les experts-comptables pour qu'ils discutent en toute confiance et trouvent des solutions : par exemple, simplifier les mesures, comme l'année blanche de cotisations sociales et bancaires. d'aides de ménage, de gardes d'enfants, afin de soutenir les femmes dont les maris vivent une période difficile, car les compagnes doivent alors prendre le relais et faire face à la multiplication des démarches administratives, tout en gérant leur travail et la famille.

Elle y décrit le bonheur d'une vie rurale, puis l'inquiétude, la dépression, le premier geste, enfin le second, qui sera fatal ... Dans ce livre, Camille se révolte, à bon droit « Tu ne t'es pas suicidé, tu as été tué, tué par tous ceux qui ont voulu profiter de toi, tué par le manque d'humanité, tué par les institutions, par tout un système qui a vu en toi un travailleur acharné créateur de richesses auxquelles tu n'as pratiquement jamais eu accès. Notre monde est devenu fou ; il tue les paysans qui l'alimentent. » Ces mots très durs nous confrontent à nos défaillances. Nous nous rendons tous coresponsables, en nous taisant, en acceptant l'inacceptable, en nous arrangeant de solutions qui ne fonctionnent pas, en ne dénonçant pas un système qui privilégie la dématérialisation et qui oublie l'humain. Le compteur tourne. Ce soir, en vous couchant, chers collègues, pensez qu'il y aura un paysan de moins,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le sujet dont nous discutons aujourd'hui est un drame qui frappe nos campagnes un jour sur deux, qui est peu documenté, peu médiatisé et qui est pourtant la manifestation la plus flagrante de la détresse du monde agricole : le suicide des agriculteurs. Je tiens à remercier notre collègue Henri Cabanel, auteur de la proposition de loi,

Seules trois études ont été réalisées sur le sujet et leurs auteurs n'ont pas suivi la même méthodologie, ce qui ne les rend pas comparables et nuit à la compréhension du problème. Pourtant, il est impossible de traiter cette problématique importante sans en avoir une bonne connaissance statistique. Une

Nous ne disposons pas de chiffres plus récents, ce qui représente un véritable obstacle à la mise en place d'une politique publique efficace. Selon cette étude, les exploitants agricoles font face à une surmortalité par suicide de 20 % par rapport au reste de la population, à trois reprises au cours des cinq années étudiées. Ces éléments démontrent déjà toute la complexité du problème. Évidemment, au-delà de ces statistiques, malheureusement froides et impersonnelles, chaque histoire est unique, singulière, avec ses drames et ses souffrances.

Les chiffres démontrent même une sous-mortalité de 20 % chez les hommes et de 57 % chez les femmes, mais avec des biais statistiques importants, comme l'exclusion des salariés-exploitants. Une troisième étude, réalisée par la MSA et publiée en juillet 2019, démontre, avec une autre méthodologie, une surmortalité par suicide des assurés du régime agricole. Centrée sur les assurés ayant reçu un soin dans l'année,

Il est absolument nécessaire que des études incontestables viennent objectiver ces éléments. Disposer de chiffres fiables est un prérequis incontournable, tant pour le législateur que pour le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'élaborer des solutions pratiques. Notre seconde Notre seconde constatation est que ce n'est pas une loi qui permettra de résoudre, une fois pour toutes, le problème du suicide des agriculteurs. Nous avons tous été confrontés, sans doute, dans nos territoires respectifs, à des cas tragiques d'agriculteurs ayant mis fin à leur jour. Ces décisions sont, le plus souvent, l'aboutissement d'une accumulation de difficultés, d'une concordance de différents drames individuels. Parmi ceux-ci figurent bien entendu les difficultés financières, mais ces dernières ne sont que la face émergée de l'iceberg. Il y a surtout les drames personnels, l'isolement social et géographique, la perte d'estime de soi, l'absence de reconnaissance, la surcharge de travail. Il y a d'autres comme les injonctions contradictoires d'une société qui a oublié que ses agriculteurs la nourrissent au quotidien, ou qui développe des fantasmes sur le prétendu subventionnement des agriculteurs, alors qu'il s'agit avant tout de la garantie de prix bas pour le consommateur. Le phénomène d'agri-bashing est en outre un facteur supplémentaire de pression sur nos agriculteurs, dans un contexte de crise de l'agriculture dans son ensemble. La loi peut être utile pour créer des dispositifs de prévention, les coordonner et les faire connaître, mais l'édiction d'une norme générale par le législateur ne permettra pas de répondre aux défis posés par ces centaines de situations individuelles. Chaque cas est singulier. Par exemple, les réactions à adopter en cas de signalement d'un agriculteur en difficulté diffèrent selon que l'alerte a été donnée par l'agriculteur lui-même, de façon volontaire, par ses proches ou par des professionnels en contact avec lui. S'il est nécessaire que la loi intervienne pour déterminer de grands principes, elle le fera, mais ce besoin n'a pas été identifié lors des auditions : les actions à mettre en place semblent, au contraire, relever du terrain, au mieux du pouvoir réglementaire. Notre troisième constatation, c'est qu'il convient de remettre l'humain au coeur des dispositifs préventifs déjà en place. Ils sont nombreux : Agri'écoute, de la mutualité sociale agricole, la MSA ; les cellules de prévention disciplinaires et les réseaux de sentinelles l'aide à la relance de l'exploitation agricole, l'ex-Agridiff. Depuis 2017, des cellules départementales d'accompagnement ont en outre été mises en place pour rassembler les principaux acteurs, en relation avec les exploitants. Enfin, de nombreux territoires ont fait le choix de solutions intéressantes, comme la Marne, avec le dispositif Réagir, qui coordonne les outils de prévention des différents organismes. Malheureusement, ces dispositifs pâtissent d'une faible lisibilité et d'une faible articulation. Il importe donc, en tout premier lieu, de faire connaître ces outils aux agriculteurs et à leurs proches. En tout état de cause, on ne peut que regretter le caractère impersonnel de ces dispositifs préventifs. Face à un homme ou une femme en détresse, c'est l'humain qui doit être au coeur de la détection et de la prévention. C'est en mobilisant les forces de chacun, dans une logique collective, et non pas individuelle, que l'on peut espérer aider les agriculteurs en difficulté. À cet égard, la présente proposition de loi présente quelques écueils. Elle crée une obligation pour une banque, en cas de déficit récurrent du compte de l'agriculteur, de l'informer de la nécessité d'alerter les organismes sociaux, puis de le faire après accord du client. Ce faisant, le salarié bancaire deviendrait le principal lanceur d'alerte, et toute la responsabilité morale pèserait sur lui. Les banques doivent, bien entendu, participer, comme tout le monde, à cet effort collectif de prévention, mais il ne paraît pas souhaitable de faire porter directement et uniquement au chargé de clientèle la responsabilité morale, voire juridique, d'un éventuel suicide de l'agriculteur. En outre, techniquement, la rédaction pose plusieurs questions, notamment dans le cas où le client serait « multi-bancarisé », ou bien dans le cas où son compte serait partagé avec son conjoint. Pour qu'un dispositif de prévention fonctionne, trois impératifs doivent être réunis : la transparence, l'effort collectif et l'humanisation des procédures. Apporter, à notre juste place, les solutions qui relèvent de notre responsabilité exige humilité et absence de précipitation. Pour toutes ces raisons, l'ensemble des membres de la commission des affaires économiques a décidé de ne pas adopter la proposition de loi en l'état,

Si vous l'adoptiez, un groupe de travail dédié à ce sujet, trop longtemps resté à l'écart du débat public, serait parallèlement créé, afin de produire un rapport faisant état de la situation et formulant les recommandations qui lui sembleraient les plus utiles. En travaillant de façon transpartisane et collégiale, nous aboutirons à un rapport de qualité et à des solutions concrètes pour améliorer les outils de prévention mis en oeuvre par l'État. Un problème aussi grave que celui-ci ne peut pas rester sans solution, et j'ai confiance dans la capacité du Sénat à réaliser un travail fin et précis, qui permette d'avancer dans la bonne direction sur ce sujet. Notre chambre représentant les territoires, notre action s'inscrit donc logiquement aux côtés de ceux qui les font vivre. Il n'y a pas de tendance qui soit irréversible ou de drame qui ne puisse être évité : nos travaux, j'en suis sûre, le prouveront. La parole

Peut-on seulement se figurer ce qui pousse un homme à mettre fin à ses jours, à trouver la vie tellement insupportable que la mort est une délivrance ? Cet acte ultime, radical, n'appartient qu'à celui qui le commet. Il faut, je pense, respecter la singularité de ce geste. Le suicide est évidemment un geste individuel, mais il a aussi des causes plus profondes, plus larges, sociales, collectives. Le père de la sociologie française, Émile Durkheim, en a fait la démonstration en 1897 dans un ouvrage fondateur,. Il y pointait les risques d'un défaut de reconnaissance et d'un délitement des liens sociaux. Je ne citerai qu'une phrase de cet ouvrage : « Le suicide varie en fonction inverse du degré d'intégration des groupes sociaux

je ne puis me résoudre, et nous ne pouvons nous résoudre ensemble à ce que des paysans de France vivent si mal leur travail que certains ne voient d'issue que la mort pour retrouver leur dignité. Le débat que vous provoquez aujourd'hui est salutaire. Plus encore, il est absolument nécessaire. Il est difficile de parler du suicide, mais nous devons le faire, dans cet hémicycle, dans les médias, au cinéma, partout, parce que cette situation ne peut être banalisée.

mais s'en servir à d'autres fins que son élimination serait manquer de respect à la mémoire de ces personnes. Ce serait inacceptable. Les derniers travaux de la MSA pour l'année 2015 confirment bien une surmortalité par suicide des assurés au régime agricole, de 15 ans à 64 ans. Cette surmortalité par rapport au régime général est estimée à 12 %.

Parmi eux, 372 exploitants et 233 salariés agricoles, pour la très grande majorité des hommes. Les taux de décès par suicide progressaient jusqu'à 40 ans, puis restaient stables, avant d'augmenter de nouveau nettement chez les plus de 65 ans. C'est plus d'un exploitant par jour qui se donnait la mort à l'époque ; ce chiffre est terrible ! Il faut admettre que nous ne connaissons pas bien les évolutions de ce drame à l'échelon national. C'est en ce sens que votre réflexion a toute sa pertinence. Certes, des études ont été réalisées, ces dernières années, et vous les avez évoquées, mais elles l'ont été avec des méthodes et des échantillons différents, donnant des résultats variables, voire contradictoires avec cette dernière étude de la MSA, ce qui ne nous permet pas d'étudier tranquillement ce qu'il en est. Les travaux que vous allez mener, dans les semaines qui viennent, avec votre commission, permettront, me semble-t-il, d'éclairer la société. Nombreux sont ceux qui avaient retenu des travaux précédents L'honnêteté m'oblige à dire qu'aucune étude ne permet de confirmer une augmentation ou une réduction du nombre de suicides dans le monde agricole ces dernières années. Il faut que nous soyons clairs sur l'ensemble de ces chiffres. C'est bien là un chantier important à mener : mieux connaître la situation et son évolution. Malgré ces difficultés à objectiver le phénomène, nombre d'autres indicateurs sont alarmants : 3 560 exploitants ont dû bénéficier d'une aide au répit en 2017 environ 300 appels sont donnés par mois au dispositif d'écoute pour les agriculteurs en situation de détresse, Agri'écoute. Les cellules pluridisciplinaires de prévention, constituées dès 2012 dans les 35 MSA, ont détecté 1 654 situations problématiques en 2018. Vous entendez chez chiffres : ils sont énormes ! Les cellules d'identification et d'accompagnement pour les agriculteurs en difficulté, mises en place par l'État dans plus de soixante-quinze départements, en sont à 2 100 signalements depuis septembre dernier. Affirmer que la faiblesse des revenus et l'endettement sont les seules causes du suicide serait, à mon sens, une simplification qui ne servirait pas notre objectif de mieux le prévenir.

Le revenu est crucial, mais il n'est évidemment pas le seul facteur. Différentes études mettent en évidence une conjonction de causes : au-delà de la pression financière et de l'endettement, il y a les problèmes interpersonnels dans la famille ou dans le groupement sociétaire, les événements particuliers de vie, les problèmes médicaux, les tracas administratifs, que vous avez évoqués, et, enfin, le temps de travail, qui est très élevé pour les agriculteurs et les éleveurs. Les études montrent aussi une forte pression sociale, qui pèse sur les agriculteurs. Il existe un sentiment de honte en situation d'endettement ou de difficulté.

Il existe une autre forme de pression, celle de l'attente sociétale, qu'a évoquée M. Cabanel, celle d'une transition des modèles agricoles et agroalimentaires. La société leur demande toujours plus, et, parfois, ils sont démunis pour répondre à ces chamboulements.

au travers du plan national de prévention. Notre action est triple : mieux connaître les données chiffrées ; proposer un dispositif d'écoute pour les agriculteurs en situation de détresse, à savoir Agri'écoute, qui est accessible à tout moment ; créer des cellules de prévention.

Il existe d'autres dispositifs d'identification : ceux de la MSA, ceux de l'association Solidarité Paysans et ceux de divers réseaux, comme le réseau Agri-sentinelles, porté par Allice et Coop de France et animé par l'Institut de l'élevage. L'État se mobilise aussi une fois que l'agriculteur en difficulté est identifié. Le ministère a développé une aide à l'audit global de l'exploitation agricole, qui vise à établir un bilan de la situation technique, économique, financière et sociale de l'exploitation. Celui-ci se fait en concertation avec l'agriculteur. Pour les difficultés économiques, une aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA), qui permet un plan de restructuration et un suivi techno-économique sur la durée, est en place.

d'y parvenir. Il nous faut également rendre plus visibles les acteurs de proximité susceptibles d'aider un agriculteur. Aujourd'hui, il y a une marge de progression assez sensible. Néanmoins, nous devons dépasser la logique de guichet et systématiser, comme certains le font, la logique de démarche vers les agriculteurs en difficulté. Nous devons aussi travailler sur le suivi des personnes ayant tenté de se suicider et améliorer l'offre de formation et la sensibilisation des acteurs. Enfin, il nous faut affiner notre compréhension sociale et nos statistiques sur la question du suicide.

le Premier ministre a souhaité confier une mission à un parlementaire sur le sujet du suicide. Elle sera soutenue par les inspections des ministères de l'agriculture et de la santé.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est un sujet particulièrement sensible que mon groupe a décidé de porter aujourd'hui dans cet hémicycle. Au détour Au détour du travail législatif que nous menons régulièrement pour le secteur agricole, nous évoquons de plus en plus systématiquement la détresse morale que vivent beaucoup d'agriculteurs et qui peut malheureusement conduire certains d'entre eux à mettre fin à leurs jours. Sur le terrain, dans nos terroirs, dans nos villages, lequel d'entre nous n'a jamais été confronté à cette tragédie humaine ? Aussi, je remercie mon collègue Henri Cabanel d'avoir formalisé cette préoccupation au travers d'une proposition de loi visant à prévenir le suicide des agriculteurs. Sans prétendre, avec ce texte, trouver dès aujourd'hui la réponse à un phénomène complexe, nous nous devons d'ouvrir ce débat pour jeter les bases d'un travail collectif autour de la question du suicide au sein du monde agricole et pour voir, ensemble, ce qui pourrait relever de notre responsabilité de législateur. Si les chiffres méritent d'être actualisés, comme l'a très justement souligné notre collègue rapporteur, les différentes études témoignent d'un phénomène alarmant, avec un taux annuel de suicide chez les exploitants qui est supérieur à celui de la population générale. Un suicide quasiment tous les jours- une réalité sans concession ! Les agriculteurs sont confrontés, dans l'exercice de leur métier, à des difficultés spécifiques indéniables, qui se cumulent négativement comme nulle part ailleurs. On le sait, le monde paysan est sans cesse sous pression. Pression des consommateurs, pression du marché, pression des distributeurs, pression des aléas climatiques, de la biodiversité et des aléas sanitaires, pression des néo-ruraux qui s'installent à la campagne campagne ; s'y ajoute plus récemment, pour les éleveurs, la pression, particulièrement agressive, d'associations antispécistes ou, pour les viticulteurs, celles des lobbies anti-alcool. Pour autant, tenaillés entre urgence économique, urgence écologique et attentes de la société, les exploitants ne ménagent pas leur peine, aujourd'hui comme hier, pour exercer la mission vitale qui leur incombe : nourrir l'humanité Souvenons-nous, après la guerre, il fallait faire de la France une grande nation agricole. À force de modernisation, les exploitants ont atteint l'objectif, au point que l'on a pu parler à l'époque de « pétrole vert Aujourd'hui, on leur demande de produire mieux et de s'engager dans la transition écologique. Là encore, la plupart d'entre eux sont au rendez-vous du défi environnemental, malgré les contraintes que cela implique en matière d'appropriation des normes et d'engagements financiers. Au bout du compte, c'est une vie d'investissement sans limites, de sacrifices personnels et, presque toujours, d'endettement, sans avoir la certitude qu'ils auront de quoi vivre. Je rappellerai que, en 2017, près de 20 % des exploitants n'avaient pu se verser de salaire, et près d'un quart d'entre eux vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Quant à la reconnaissance de la société, elle se mesure à l'aune de ce mot barbare, mais si parlant : l'agri-bashing. Il est de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme : une société qui ne respecte plus ses agriculteurs et qui n'est plus en mesure d'assurer son indépendance alimentaire est une société en perdition. Cette proposition de loi vise à créer une alerte par l'intermédiaire des banques, en fonction de la situation financière des exploitants. Certes, cela n'est pas suffisant pour appréhender toutes les situations. Toutefois, mon collègue Henri Cabanel l'a souligné, les services du ministère de l'agriculture ont observé un lien prépondérant entre endettement et suicide. Soyons clairs, ce texte est, à ce stade, un appel, qui est urgent. Il doit permettre, je l'espère, monsieur le ministre, d'apporter rapidement des réponses, que celles-ci soient nouvelles ou généralisent les dispositifs qui existent- vous les avez rappelés -, mais qui sont si souvent méconnus. défaut, le retour de manivelle sera encore plus violent. En attendant un examen du texte plus poussé en commission, il est indispensable de poursuivre au Sénat notre travail plus général de soutien au monde agricole, ce qui revient à s'attaquer aussi aux causes profondes des situations de détresse. Comme je l'ai déjà indiqué, il est essentiel d'accompagner les mutations demandées au secteur, pour que celles-ci soient économiquement supportables. À cet égard, nous attendons avec impatience l'évaluation de la loi Égalim, en particulier de ses dispositions censées améliorer les revenus des agriculteurs. Il faut également se battre pour maintenir les moyens de la PAC, Je pense aussi à l'assurance récolte, qu'il serait souhaitable d'améliorer, comme le souligne la proposition de résolution sur ce sujet que j'ai déposée avec mes collègues Yvon Collin et Henri Cabanel. au-delà du soutien que l'on doit porter à l'activité, je n'oublie pas ce qu'il nous faudra faire pour rompre la solitude dans laquelle sont plongés des milliers d'hommes et de femmes sur nos territoires, rompre l'isolement du monde rural, de « ces hautes terres où la solitude a rouillé l'herbe » pour reprendre quelques mots de Jean Giono. Cela passe par le maintien des services publics auprès de ces hommes et de ces femmes, qui sont eux-mêmes, par leur présence sur leur terre et par leurs activités, de puissants acteurs de l'aménagement du territoire. N'oublions pas cette réalité et rappelons simplement et rappelons simplement à tous nos concitoyens que les agriculteurs sont les garants de nos vies. La parole

Nous avons tous en tête ce chiffre terrible : un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Je voudrais en premier lieu remercier notre collègue, Henri Cabanel, d'avoir porté cette proposition de loi, qui nous permet aujourd'hui d'aborder ce sujet si délicat au sein de notre hémicycle. Pendant des années, cette détresse des agriculteurs a été occultée, comme un tabou dans notre société. Il a fallu attendre 2011 pour que l'État, avec la MSA, s'engage sur cette question. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a été chargée par Bruno Le Maire, alors ministre de l'agriculture, de mettre en oeuvre un programme national d'actions, afin de recueillir des données chiffrées sur la réalité du suicide chez les exploitants et les salariés agricoles. Répondre aux alertes, accompagner, orienter et suivre ces personnes en détresse : tels sont les axes qu'il faut suivre Toutefois, il est impossible de prétendre traiter cette problématique sans avoir une bonne connaissance des différentes dynamiques qui mènent un individu à des pensées noires et qui le poussent à passer à l'acte. Certes, nous pouvons présumer que ces drames sont intimement liés à la situation financière du défunt. En effet, on observe une proportion bien plus grande de suicides d'agriculteurs dans les filières les moins rémunératrices ou durant les périodes où les prix de vente de ces mêmes filières sont les plus bas. Je pense tout particulièrement aux éleveurs bovins laitiers et allaitants.

Les agriculteurs font face aux risques économiques de leur métier, au surendettement, mais aussi aux aléas de la vie, comme la solitude ou la maladie. La pression exercée sur eux est aussi un facteur à prendre en considération. Nous ne le répéterons jamais assez : il faut que l'agri-bashing cesse Cette proposition de loi entend apporter une solution de prévention pour éviter ces suicides. Elle vise à améliorer le système de détection des personnes en situation de fragilité dans le monde agricole, en instaurant un repérage ciblé des personnes à risque en fonction de leur niveau d'endettement ou de leurs difficultés financières et en plaçant les établissements bancaires au coeur du dispositif d'alerte. Ces derniers sont Sensibiliser les banques sur cette question en les obligeant à repérer les difficultés d'un client agriculteur et à l'orienter vers un accompagnement social et psychologique est une mesure de bon sens. Elle rejoint l'action menée par le Gouvernement dans la prévention du risque psychosocial et de l'épuisement professionnel ; monsieur le ministre, je connais votre engagement en la L'instauration d'une visite médicale annuelle pour les agriculteurs avec un médecin du travail est également une bonne chose. Elle doit faire l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux concernés. Nous savons que ces drames ont des causes multiples. Toutefois, ne nous leurrons pas : si nous nous préoccupons aujourd'hui de la dimension financière, bien qu'elle ne doive pas être dissociée du reste,

En vérité, mes chers collègues, aucune loi ne permettra de résoudre, une fois pour toutes, le problème du suicide en général, et celui des agriculteurs en particulier. C'est pour cette raison que je rejoins l'avis de Mme le rapporteur : nous devons prendre le temps de mieux étudier et de comprendre ce phénomène- j'irai plus loin, ce désastre -dans toute sa complexité, d'explorer l'ensemble des pistes et d'apporter, autant que possible, des idées permettant d'améliorer la prévention. Le groupe La République En Marche votera donc la motion de renvoi à la commission,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, évoquer, échanger et débattre sur le suicide, en particulier sur celui des agriculteurs, suppose un débat exigeant et sérieux, pour apporter

Se suicider, mettre fin à sa vie, c'est l'un des gestes les plus terribles qui soient. Il n'y a pas une seule cause ; elles sont multiples : rupture, maladie, isolement, problèmes personnels, financiers ou professionnels, etc. Prévenir les suicides demande donc de prendre l'ensemble de ces facteurs en compte et de tenter d'y apporter une réponse globale, mais adaptée à chacune et à chacun. C'est pour cela que nous partageons l'avis de la commission et de l'auteur de la proposition de loi, Henri Cabanel- je tiens d'ailleurs à le remercier sincèrement de son travail

Le monde paysan a été confronté à des changements radicaux depuis la fin des années 1960 : mécanisation, impératifs d'augmentation de la productivité, utilisation de nouveaux pesticides, perte d'autonomie sur les semences, informatisation, charges administratives et comptables toujours plus importantes. Bref, nos agriculteurs font face à un changement permanent. Or toutes ces adaptations ont eu pour conséquence ce que l'on a appelé « l'endettement obligé pour s'inscrire dans la modernité ... -et la pression de plus en plus grande de cet endettement sur la vie quotidienne. Tout cela dans un contexte de libéralisation croissante des échanges et des marchés et de pression des agro-industriels et de la grande distribution. Sans compter la volonté de multiplier encore et toujours les accords de libre-échange qui sont et seront les fossoyeurs du modèle agricole familial que nous défendons Que dire encore de l'envolée des prix du foncier et de la défiance que suscite cette profession parmi une population qui ne veut plus de pesticides, qui refuse la malbouffe et qui est de plus en plus sensible aux scandales sanitaires et environnementaux, souvent à raison ? Ainsi, les agriculteurs sont pris en tenaille. D'un côté, il y a les remboursements des emprunts et le coût exorbitant des produits et pesticides, qui s'accompagne d'une sorte de captivité des agriculteurs face aux entreprises « phyto », comme nous avions pu le dénoncer lors de l'examen De l'autre, il y a les prix tirés vers le bas par la grande distribution, prix qui ne permettent plus de vivre décemment. Il est insupportable de se dire que, aujourd'hui, ces hommes et femmes qui nous nourrissent vendent leurs productions à perte et n'arrivent même pas à se payer un SMIC, alors qu'ils travaillent sept jours sur sept, plus de dix heures par jour. Tout cela pour subir finalement un niveau de retraite indécent après une longue vie de dur labeur. À cet égard, et sans polémiquer,

Comment ne pas rappeler qu'il s'agissait alors, comme aujourd'hui, de répondre à une urgence sociale, celle des retraités agricoles qui ne peuvent pas vivre dignement ? En effet, comment parler de dignité quand le niveau de revenu se situe entre 700 et 800 euros en métropole et se réduit parfois à seulement 100 euros dans nos territoires ultramarins ? Comment peut-on vivre avec moins que le seuil de pauvreté et que le minimum vieillesse ?

notre souveraineté alimentaires. Je rappelle ces éléments, car c'est en les prenant tous en compte que nous pourrons travailler efficacement ensemble à prévenir les suicides dans le monde agricole. Enfin, nos agricultrices et agriculteurs vivent dans ce que l'on appelle les zones blanches. Alors que toutes les politiques accélèrent la métropolisation, en concentrant les lieux de pouvoir, de savoir et d'activités économiques, ceux qui vivent en ruralité ont l'impression d'être abandonnés. Les écoles ferment, les services publics fuient les uns après les autres, les centres-bourgs se dévitalisent et l'essence qui est nécessaire pour se déplacer- il n'existe aucun transport public de plus en plus cher. Quand il faut mettre une heure de voiture pour se rendre en ville ou aller se faire soigner ou qu'il faut parcourir plus de 25 kilomètres pour aller chercher une baguette de pain, le sentiment d'abandon et d'injustice est renforcé. C'est donc, là aussi, les politiques d'austérité publique qu'il faut questionner et l'égalité territoriale qu'il faut exiger pour nos territoires ruraux, au même titre que pour nos quartiers populaires et nos territoires ultramarins. Les gouvernements successifs portent la responsabilité de cette souffrance sociale, et le vôtre, malgré les promesses de la loi Égalim, n'a rien fait, bien au contraire, pour enrayer cette spirale mortifère. Nous pensons donc que le mécanisme d'alerte proposé par la proposition de loi ne règlera pas seul le problème, mais je suis certain que

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, on compte plus d'un suicide par jour chez les agriculteurs. Les chiffres sont alarmants, et la réalité est encore plus sinistre. C'est pourquoi je tiens à saluer et à remercier le groupe RDSE, en particulier notre collègue Henri Cabanel, qui a mis ce sujet dramatique et bouleversant au coeur de l'agenda de notre assemblée des territoires. Comme l'a si bien rappelé Mme le rapporteur en commission la semaine dernière, ce sujet révèle « la manifestation la plus flagrante de la détresse du monde agricole Force est de constater que ce fléau qui touche nos territoires ruraux est malheureusement plus présent dans le monde agricole que dans d'autres secteurs d'activité. Les causes de ce phénomène dramatique sont multiples : difficultés financières, drames personnels, maladie, isolement social et territorial, surcharge de travail, agri-bashing, aléas climatiques, manque de visibilité sur l'avenir. Ces situations irrémédiables sont le plus souvent le fruit d'une accumulation de difficultés et de la concordance de drames personnels de toute nature, même si le contexte économique est sans doute déterminant. Ce phénomène touche toutes les tranches d'âge, les jeunes comme les moins jeunes, tous les métiers du secteur, les salariés et les exploitants. Les chiffres sont clairs, ils parlent d'eux-mêmes et sont glaçants la MSA relève 605 décès par suicide par an dans le milieu agricole, exploitants et salariés confondus, parmi lesquels 274 avaient plus de 65 ans

De plus, deux activités sont particulièrement concernées : les éleveurs bovins et les producteurs laitiers. En France, les agriculteurs ont un risque de suicide plus élevé de 12 % comparé au reste de la population.

De multiples leviers doivent donc être actionnés, afin de proposer une solution concrète et complète aux agriculteurs de notre pays. Je pense d'ailleurs que les actions les plus efficaces à mettre en place relèvent du terrain. Il est néanmoins impératif que ces initiatives fassent l'objet de davantage de visibilité : force est de constater que, aujourd'hui, les dispositifs locaux sont encore trop mal connus, ce qui est dommageable pour leur efficacité. Dans mon département, la Meuse, la chambre d'agriculture a mis en place un numéro vert Ce dispositif permet une orientation vers des personnes formées et des entités compétentes en fonction des besoins, qu'ils soient économiques, de santé ou autres. Le travail d'accompagnement se fait ensuite en coopération avec les acteurs en présence- la chambre d'agriculture, la MSA,

ont instauré des processus similaires dès les années 2000. Un guichet unique a été créé en 2018 ; il est accompagné d'initiatives qui ont prouvé leur efficacité : aide financière au soutien psychologique, aide pour la comptabilité ou encore aide au répit. force est de constater que les signaux d'alerte se déclenchent souvent trop tard. La détection est certes complexe, et des pistes d'amélioration du dispositif d'accompagnement sont à trouver. Aussi, il est nécessaire d'identifier, d'une part, les initiatives locales efficaces et, d'autre part, les secteurs en besoin. Je crois que la coordination et la formation des acteurs sont indispensables pour anticiper et identifier les signes précurseurs. À mon sens, une adaptation territoriale est donc un axe de réflexion à approfondir. L'aide L'aide doit être plus globale et inclure des volets financier, économique, social et technique, ainsi qu'un accompagnement plus individualisé. Il faut remettre de l'humain dans un dispositif qui, souvent, est trop impersonnel. En résumé, il est nécessaire d'anticiper les risques

avant d'entrer dans l'analyse de cette proposition de loi, je voudrais tout d'abord remercier notre collègue Henri Cabanel, qui nous donne l'occasion de consacrer une séance publique de la Haute Assemblée à cette terrible réalité qu'est la surmortalité par suicide des agriculteurs. Les chiffres sont alarmants : la récente étude de la MSA fait état de 605 décès par suicide en 2015, dont 372 chefs d'exploitation- 292 hommes et 80 femmes, soit un suicide par jour environ -et 233 salariés agricoles.

Ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis la fin des années 1960 et l'apparition des données de suicide par catégories socioprofessionnelles, on constate que les agriculteurs sont au sommet de la pyramide des suicides. Toutefois, pendant longtemps ces données sont restées dans l'ombre. Comme dans le reste de la société, le suicide est un tabou dans le monde agricole, et peut-être plus encore, car, au-delà de la honte associée à ce décès, le suicide a souvent été exclu des garanties des assurances. Aussi, des générations de paysans ont tu les suicides de leurs collègues, les faisant passer pour des accidents. Cette problématique a commencé à percer dans le débat public au moment de la crise du lait en 2009. Aujourd'hui encore, les éleveurs bovins et les producteurs laitiers sont particulièrement touchés. Le film, sorti il y a quelques mois, a également contribué à mettre en lumière ce fait social majeur. Nous avons eu la chance de pouvoir assister à une projection-débat la semaine dernière au Sénat, en présence de l'équipe du film. Pour celles et ceux qui, comme moi, vivent ou ont vécu du travail de la terre, il sonne de manière très juste- si juste qu'il peut être extrêmement douloureux à regarder jusqu'à la fin. Aujourd'hui, grâce à la proposition de loi de notre collègue Henri Cabanel, nous disposons d'un temps dédié dans cet hémicycle pour aborder les réponses que nous pourrions apporter en tant que législateurs. Dès lors que nous n'acceptons pas le suicide comme une fatalité, la première de ces réponses est nécessairement la prévention. Le professeur Michel Debout, précurseur en France de l'approche en santé publique du suicide, plaide depuis longtemps en faveur d'une politique de prévention rénovée et renforcée, qui permettrait, comme dans d'autres pays, d'éviter de nombreux suicides. Avec ce texte, notre collègue nous propose une piste pour contribuer à la détection des paysans en détresse : faire des agents bancaires des acteurs de cette prévention. Ainsi, ces agents qui repéreraient des signaux faibles financiers auraient la possibilité de signaler leurs clients agriculteurs en difficulté financière, avec leur accord exprès, à une structure de suivi et d'écoute de la MSA. Si l'intention est incontestablement louable, les indicateurs, les outils de suivi et les acteurs responsabilisés dans cette proposition de loi ont été sérieusement mis en question tout au long des auditions que nous avons conduites ces dernières semaines. Face à un fait social aussi complexe et multifactoriel que le suicide, une réponse aussi parcellaire ne peut bien évidemment pas être adéquate. Il nous semble que d'autres pistes pourraient être utilement explorées pour améliorer la détection et la prévention des passages à l'acte. Au-delà, il nous paraît fondamental de pouvoir intervenir à un niveau structurel pour lutter efficacement contre le suicide des agriculteurs. Le « sursuicide » dans le monde agricole résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs. La situation économique des agriculteurs ou leur surendettement n'explique pas à eux seuls la dépression profonde qui conduit au suicide. À cette détresse économique s'ajoutent d'autres grands facteurs de risques : l'isolement social, une intrication tout à fait particulière entre vie familiale et vie professionnelle, l'effondrement du sens donné à sa vie face à l'impossibilité de transmettre l'exploitation, ce qui explique notamment la proportion importante de suicides chez les agriculteurs âgés, ou encore la perte brutale de repères ou de perspectives lors de la survenue d'événements climatiques lourds, par exemple. Le paysan ne partage pas facilement ses difficultés avec son voisin ou même sa famille. Le fera-t-il plus facilement avec le gestionnaire de son compte en banque ? C'est pour ces raisons que les membres du groupe socialiste et républicain estiment qu'un employé de banque n'est pas forcément le mieux placé ou formé pour aider un agriculteur en difficulté. Comment un agent bancaire sans formation saura-t-il trouver les bons mots pour proposer à son client de le signaler à la MSA ? C'est une responsabilité bien lourde à confier à des personnes qui n'ont reçu aucune indication dans leur formation initiale pour intervenir de manière appropriée auprès de personnes particulièrement fragiles. En outre, de par sa profession, l'employé de banque ne peut apprécier que la variable économique. Or être à découvert fait partie intégrante de la vie des agriculteurs ! Cet indicateur nous apparaît donc comme peu pertinent. De même, les auditions ont fait ressortir que l'anonymat était l'un des facteurs permettant la réussite du système d'écoute proposé par la MSA. Un tel mécanisme mettrait nécessairement à mal ce préalable de l'anonymat pour un bénéfice difficile à appréhender en l'état. Cependant, nous souhaiterions que d'autres pistes de réflexion puissent être explorées, pour enrichir le travail de notre collègue Cabanel. Ainsi, d'autres lanceurs d'alerte pourraient être mis à contribution, parmi ceux qui sont au contact direct des paysans. Il pourrait s'agir des vétérinaires, des coopératives agricoles, des syndicats, des chambres d'agriculture ou encore des travailleurs sociaux. Édouard Bergeon, le réalisateur du film, appelle à soutenir davantage l'association Solidarité Paysans, dont les équipes accompagnent depuis plus de trente ans les agriculteurs en difficulté dans nos territoires. Elles ont la connaissance des mécanismes à l'oeuvre et le savoir-faire pour y répondre, elles disposent sont loin d'être à la hauteur des enjeux. Il pourrait également être intéressant de travailler sur des pistes ciblant précisément certains des facteurs de risques recensés, par exemple lutter contre l'isolement social dans nos campagnes- même aujourd'hui, au XXI siècle, on se suicide quatre fois plus en milieu rural qu'à Paris organiser un meilleur accompagnement des agriculteurs victimes des aléas climatiques. Cependant, nous n'aurons fait que la moitié du chemin tant que nous ne nous serons pas penchés sur les causes profondes de cette surexposition des agriculteurs au risque de suicide. Le modèle productiviste actuel actuel entraîne nos paysans dans une spirale de crédits et de factures à payer. Ils subissent ainsi la surenchère du « toujours plus grand », qu'il s'agisse des augmentations de rendement, des volumes de prêts bancaires contractés, des surfaces à cultiver, du nombre de bêtes à élever ... Ce « toujours plus » crée un véritable cercle vicieux, qui entre en résonnance avec les autres problématiques des agriculteurs. Or cette spirale financière et économique entraîne également l'épuisement moral et physique. En effet, si les surfaces et les nombres de têtes croissent, les bras manquent, tandis que les factures et les dettes s'accumulent. Contrairement à ce qui est martelé, ce n'est pas l'agri-bashing qui pousse les paysans au suicide, mais le modèle d'agriculture productiviste. Aussi, l'évolution du modèle agricole vers un mode de production raisonné et raisonnable permettrait de préserver non seulement notre planète, mais aussi le bien-être au travail de nos agriculteurs. Cette proposition de loi permet donc de mettre la question du suicide des paysans à l'ordre du jour de nos travaux. Elle offre l'occasion de mener un véritable travail parlementaire. Cependant, le texte tel qu'il a été écrit ne permet pas d'embrasser l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et structurels, qui sont au coeur du mal-être des paysans. En tant que parlementaires, nous devons construire un système plus complet de réponses à ce fait social inacceptable : ceux qui nous nourrissent ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail et de plus en plus de raisons d'en mourir. C'est pour cela que le groupe socialiste et républicain votera la motion de renvoi à la commission.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Jean Giono, grand poète de la terre et des paysans, disait que « l'essentiel n'est pas de vivre, mais d'avoir une raison de vivre Cette raison de vivre, de trop nombreux agriculteurs français semblent l'avoir perdue. Chaque année, des centaines d'entre eux commettent l'irréparable. Tous les jours, un agriculteur se suicide en France ; un chiffre glaçant, qui souligne l'urgence d'agir pour prévenir le suicide dans le secteur agricole. Les raisons du malaise paysan sont aussi profondes que multiples. Les causes les plus visibles sont souvent d'ordre financier. C'est cet axe qu'a choisi notre collègue Henri Cabanel pour proposer une réponse pragmatique et parer à l'urgence. Ne nous voilons pas la face ! La question des revenus agricoles est majeure et notre modèle économique agricole français nécessite d'être repensé en profondeur. Trop peu d'agriculteurs vivent décemment du fruit de leur travail.

Cette réalité, je la connais pour être né dans une ferme et avoir exercé le beau métier d'agriculteur-éleveur pendant plus de quarante ans. Au long de ces années, j'ai vu le système changer et prendre au piège les agriculteurs français.

sur des surfaces toujours plus grandes, et souvent en monoculture. Ce gigantisme et cette course à la productivité ont obligé certains agriculteurs à s'endetter et à entrer dans la spirale du « marche ou crève À cela est venue s'ajouter la politique agricole commune, une bonne idée qui s'est peu à peu transformée en un cercle vicieux. Il est indispensable de le rappeler à l'origine, la PAC était conçue pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à des produits agricoles de qualité et à bas coûts. Aujourd'hui, le système s'est transformé en une épée de Damoclès pour nombre de nos agriculteurs, pris en tenaille entre une exigence de qualité très élevée et une guerre des prix intenable. La question financière ne touche pas que les agriculteurs actifs. Elle concerne également les travailleurs agricoles au chômage et les retraités. Dans cet hémicycle, j'ai interpellé le Gouvernement, comme beaucoup d'autres de mes collègues, sur la question de l'assurance chômage des agriculteurs. La seule réponse a été : « Plus tard ». Même réponse pour les petites retraites. Mais plus tard, c'est trop tard ! Combien de nos agriculteurs touchent à peine 400 euros de retraite par mois ? Même pas l'équivalent du RSA pour toute une vie de travail et d'efforts. C'est inacceptable À cela s'ajoute un autre sujet, trop peu évoqué, celui des agricultrices sans statut, qui ont travaillé aux côtés de leur mari exploitant agricole et qui ne touchent aucune retraite. Tous ces sujets méritent d'être enfin considérés comme une priorité, pour faire évoluer les revenus de nos agriculteurs et offrir des garanties économiques à la hauteur du travail fourni. Cependant, la question financière est loin d'être la seule à alimenter le malaise paysan. Le sujet de la transmission me semble également central. Avoir travaillé toute une vie sans parvenir à passer le relais et revendre son affaire peut être vécu comme un véritable échec professionnel et personnel. Qu'il s'agisse du refus des descendants de poursuivre l'activité agricole ou de l'absence de repreneurs motivés, les difficultés de transmission nourrissent la souffrance psychologique. Nombre de nos agriculteurs éprouvent un sentiment d'isolement, voire de marginalisation. Travailler sans relâche, ne s'autoriser ni vacances ni loisirs ou à peine, voir le fruit de son travail ruiné en quelques minutes par une inondation, le gel ou la sécheresse, tout cela peut créer beaucoup de frustrations et une impression de déconnexion avec une société de plus en plus tournée vers le loisir et le confort au travail. Cette frustration se transforme en colère quand l'agri-bashing devient une mode.

qui prennent tout sur leurs épaules. Dans mon département de Loir-et-Cher, l'adage dit : « Petit causeux, grand faiseux. » Il est précisément temps de libérer la parole et de changer les mentalités Il faudrait également évoquer le poids des normes et des charges, ainsi que la concurrence faussée entre nos paysans français et les producteurs d'autres pays, soumis à des normes moins strictes. Le sentiment d'injustice que ressentent beaucoup d'agriculteurs ne peut que renforcer leur impression d'être déconsidérés, voire méprisés. Mon but est non pas d'établir un inventaire à la Prévert des raisons de ce malaise, mais de partager mon expérience en tant qu'ancien éleveur et élu de terrain, terrain, afin d'alimenter la réflexion que nous engageons, ensemble, aujourd'hui. La proposition de loi de notre collègue Henri Cabanel est un point de départ indispensable pour, enfin, avancer sur ce sujet.

Avec l'esprit de dialogue et d'ouverture qui est le sien, le Sénat saura poser les bonnes questions et, je l'espère, apporter des réponses à la hauteur de cet enjeu majeur Je conclurai mon propos en soulignant que la détection des situations de détresse et la prévention du suicide des agriculteurs doivent s'accompagner d'un suivi sur le long terme. Accompagner nos agriculteurs, c'est aussi les aider à se reconstruire, mais aussi, parfois, à se reconvertir et à dessiner des perspectives d'avenir motivantes. Ce ne sera possible qu'en brisant l'isolement de nos paysans et en unissant les forces et les compétences du plus grand nombre. L'agriculture est notre bien commun ! La parole est à Mme

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le chiffre fait froid dans le dos : tous les deux jours, en France, un agriculteur met fin à ses jours. Derrière ce geste irréparable, il y a parfois, à l'évidence, des raisons personnelles, mais il y a toujours le malaise qui ronge depuis plusieurs années l'agriculture française. Le monde paysan va mal ! Les difficultés financières et les problèmes de trésorerie touchent aujourd'hui toutes les filières, ou presque. Le revenu moyen des agriculteurs est nettement inférieur au SMIC, pour une moyenne de 54 heures travaillées par semaine. Et combien d'entre eux vivent au-dessous du seuil de pauvreté ? Le suicide est souvent l'acte ultime d'un homme ou d'une femme qui a tout tenté pour sauver son exploitation, en vain. À ce sentiment d'échec peuvent s'ajouter l'isolement social, la surcharge de travail, mais aussi le phénomène de l'agri-bashing, véritable guerre d'usure psychologique contre le monde agricole. Cette pression supplémentaire sur la profession est d'autant plus insupportable que certains médias semblent davantage prêter attention aux pratiques totalitaires de certaines associations qu'aux graves difficultés des agriculteurs. Comment comprendre que, un jour de tempête de neige, ils soient considérés comme des héros pour, les premiers, avoir dégagé nos routes, et que, le lendemain, ils soient montrés du doigt, pour ne pas dire jetés en pâture, lorsqu'un problème sanitaire ou environnemental resurgit dans le débat public ? ? Pourtant, quel autre secteur d'activité a réussi, en à peine vingt ans, à réaliser autant d'efforts et à bouleverser autant ses pratiques pour réduire son empreinte écologique ? Si notre pays a une longue tradition agricole, il semble aujourd'hui avoir l'agriculture honteuse.

abandonnés, ensuite, par le Gouvernement, qui, malgré des États généraux de l'alimentation lancés en grande pompe, n'a toujours pas réglé la question des marges et des revenus agricoles. Nos agriculteurs n'en peuvent plus des discours officiels de fausse compassion et des opérations de communication. Ce qu'ils attendent, ce sont des actes forts et réels Ils attendent l'arrêt de l'inflation de normes déconnectées des réalités du terrain. Ils attendent un gouvernement qui les défend à l'échelon européen et qui se bat pour redonner une préférence claire à nos produits agricoles. La proposition de loi de notre collègue Henri Cabanel a le mérite d'ouvrir le débat sur le suicide des agriculteurs. Je l'en remercie sincèrement. Le système de signalement qu'il propose est intéressant, dans la mesure où il vise à améliorer l'assistance humaine apportée aux agriculteurs.

Ajoutons que le suicide d'un agriculteur signifie souvent, à terme, la fin d'une exploitation agricole dans laquelle sa famille s'était investie depuis plusieurs générations. Pensons aux difficultés que rencontre la veuve de l'agriculteur pour reprendre l'exploitation et la transmettre à ses enfants ! À la souffrance du deuil s'ajoute la solitude face à une administration qui est souvent aux abonnés absents. La longueur des procédures- parfois plus d'un an -pénalise les familles lorsqu'il s'agit, par exemple, de débloquer les comptes, ou encore d'obtenir une décision du juge des tutelles pour l'avenir des enfants. les solutions à apporter, soyons réalistes : une loi seule ne permettra pas de résoudre définitivement ce problème. Le sujet est si vaste, si complexe ! Voilà pourquoi, comme vous, madame le rapporteur, j'estime qu'il est sage de renvoyer ce texte à la commission. Ne pas adopter ce texte aujourd'hui ne signifie pas que nous nous désintéressions du sujet. Bien sûr ! Bien au contraire, nous estimons que la gravité du phénomène oblige à élargir la réflexion et à prendre le temps qui s'impose pour en appréhender la complexité et apporter les meilleures solutions. Nous pourrions d'ailleurs élargir la réflexion aux chefs d'entreprise, qui connaissent eux aussi un taux de suicide élevé, phénomène que j'avais mesuré avec notre collègue Stéphane Artano lorsque nous avions rédigé notre rapport sur la santé au travail. Mes chers collègues, on a longtemps cru que la ruralité protégeait du suicide et que la souffrance au travail était un problème des villes. Ce n'est plus vrai ! Chaque suicide d'agriculteur est un cri de désespoir qu'il faut entendre. Ce sujet doit mobiliser l'ensemble de la communauté nationale, parce que nous sommes tous concernés. Si l'on veut encore manger demain des produits sains, qui ne viennent pas de l'autre bout du monde, nous avons besoin de nos agriculteurs. Leur bien-être au travail doit donc doit donc être une préoccupation majeure. Je me réjouis que le Sénat, par cette proposition de loi, montre une nouvelle fois la voie à suivre. Qui n'a jamais eu à connaître de près un suicide doit du moins comprendre la détresse de la personne et de sa famille :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à prévenir le suicide des agriculteurs. D'emblée, je tiens à exprimer mon soutien à ce texte, bien qu'il soit, reconnaissons-le, une bien modeste réponse face à l'ampleur du mal que nous avons pour ambition de combattre. Oui, mes chers collègues, il est temps de nous réveiller ! Réveillons-nous face à la souffrance que connaissent nos agriculteurs depuis tant d'années, depuis trop d'années maintenant. Je sais que, tous autant que nous sommes, élus des territoires, nous connaissons la beauté et l'importance du travail de nos agriculteurs, qui, chaque jour, permettent aux Français de remplir leurs assiettes de produits de qualité. Si la France est un pays qui a la chance d'être indépendant dans sa production agricole, autonome dans sa consommation et, surtout, reconnu à travers le monde pour la qualité de ses produits, c'est parce que des hommes et femmes d'exception exercent ce métier, parfois au prix de leur vie. Nous avons plus que jamais le devoir de répondre à une souffrance qui conduit parfois à commettre l'irréparable, une souffrance profonde, qui touche la plupart de nos agriculteurs. Cette souffrance puise ses causes dans de nombreux facteurs ; ce sont eux que nous devons combattre pour endiguer les maux que nous souhaitons voir disparaître. Le suicide chez nos agriculteurs n'est pas une fatalité. S'il est des exploitations qui prospèrent, ce dont nous nous réjouissons, d'autres subissent un préjudice dont

Or comment faire quand l'on reçoit moins du produit que l'on vend que ce qu'il a coûté à produire ? On ne fait pas, on subit ! On est obligé d'emprunter, de s'endetter en espérant des lendemains meilleurs. Ce modèle économique n'est aucunement supportable.

pression administrative et de contrôle, pression sanitaire et normative, pression financière et fiscale- le mal français en général. Comment ferions-nous, à la place de nos agriculteurs, pour gérer leur entreprise dans de telles conditions sans subir les conséquences physiques et psychologiques que tout cela implique ? ? Comme si cela n'était encore pas suffisant, comme si notre propre modèle n'était pas déjà suffisamment contraignant et nocif pour nos agriculteurs, nous les jetons dans la broyeuse mondiale de la concurrence déloyale.

il y va de notre responsabilité collective. Ainsi, nous en finirons avec l'agri-bashing ambiant, qui fait constamment peser la suspicion sur les agriculteurs.

À l'époque où les consommateurs veulent bien manger, mieux manger, il faut saisir cette occasion de privilégier la consommation locale, que ce soit au travers des circuits courts ou de la grande distribution. Surtout, attaquons-nous enfin aux racines du mal qui pousse chaque année tant de nos paysans à se donner la mort. C'est ainsi seulement que nous parviendrons réellement à éradiquer ce fléau.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le silence qui règne au sujet du suicide des agriculteurs doit être brisé ; nous l'avons entendu dire sur toutes les travées de notre hémicycle. L'occasion nous est donnée de le faire dans cette chambre. à remercier de nouveau notre collègue Henri Cabanel pour son initiative importante. Monsieur le ministre, vos propos ont été forts et nous ont touchés. Je veux croire que nous pouvons compter sur vous ; c'est ce que j'ai compris de vos paroles. Ainsi que je l'ai déjà souligné, le suicide d'un agriculteur est l'aboutissement d'une accumulation complexe de facteurs, d'un ensemble de pressions, de drames, de craintes, d'injonctions contradictoires et de sentiments de déconnexion, l'absence de reconnaissance morale et financière. Il y a autant de causes qu'il y a de décès, ce qui limite d'autant la possibilité de légiférer sur le sujet. En outre, la connaissance même de cette problématique n'est pas assurée. Trop peu d'études ont été réalisées ; leurs conclusions sont souvent divergentes. Nous ne pouvons pas édicter de normes

Une loi risquerait, au mieux, de n'aborder qu'une petite partie du problème et, au pire, de se révéler inapplicable sur le terrain et de susciter beaucoup de déception. Il faut donc commencer par mieux connaître et comprendre ce phénomène ; nous en sommes d'accord. Certes, des dispositifs d'identification et de prévention existent, mais ils sont bien souvent peu coordonnés entre eux, quand ils le sont même. Ils sont aussi souvent mal connus des agriculteurs et de leurs proches. Des marges de progression existent donc en la matière ; on devra notamment accorder impérativement une place centrale à l'humanisation des procédures. N'oublions pas qu'un agriculteur qui commet l'irréparable est un agriculteur qui se sent profondément seul

C'est pour se donner ce temps nécessaire que la commission des affaires économiques vous propose, mes chers collègues, cette motion. Si elle est adoptée, notre commission créera dans la foulée un groupe de travail transpartisan sur les moyens mis en oeuvre par l'État en matière de prévention,

Travailler sur ce sujet dans toute sa complexité, de façon transpartisane et collégiale, permettra d'aboutir, j'en suis sûre, à un rapport de qualité qui proposera des solutions concrètes.

où se mélangent des aspects intimes, personnels et profondément humains, et des questions de politique globale qui portent sur notre modèle agricole et commercial. Il est donc important que le Sénat se penche de manière approfondie sur cette question. Je voudrais à mon tour saluer notre collègue Henri Cabanel

véritablement finalisé, il n'en est pas moins important, car il permet d'amorcer un travail, de lancer l'alerte sur ce sujet sensible et, surtout, de briser le tabou qui l'entoure encore trop souvent. Il sera également important de replacer cette thématique dans une réflexion plus globale sur le modèle agricole. Comment rémunérer les agriculteurs au prix juste et rééquilibrer leur rapport de force inégal avec l'industrie agroalimentaire et la grande distribution ? Comment maintenir le budget de la PAC et faire en sorte qu'il soit réparti de façon plus juste entre les agriculteurs ? Comment accompagner les agriculteurs les moyens de faire évoluer leurs pratiques afin d'aller vers des modèles de production plus résilients, plus rémunérateurs, plus vertueux et plus en phase avec les attentes de la société ? Comment améliorer les relations des agriculteurs avec les institutions, en particulier dans des situations humaines complexes

potentiellement exposés à des risques de suicide. Ces acteurs souffrent pourtant trop souvent d'un manque de moyens, et cela bien que l'essentiel de leur activité soit exercé par des paysans bénévoles, le plus souvent retraités. Le lien humain et la solidarité rurale sont essentiels

du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et prorogeant le mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (procédure accélérée